La séance est ouverte.

madame la rapporteure générale,

au mépris de l'intégrité et de la souveraineté de ce pays et en rayant totalement les accords de Minsk. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite condamner avec la plus grande solennité cet acte de guerre intolérable, qui met en péril la sécurité de notre continent, et exprimer notre solidarité au peuple ukrainien injustement agressé.

j'ai vu tous les drapeaux européens, synonymes d'une paix retrouvée après les terribles événements de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la paix en Europe et la paix dans le monde sont menacées.

le comité de liaison parlementaire initialement prévu demain après-midi, car il me semble indispensable de le réunir dans les meilleurs délais. De la même manière, en écho à la proposition faite ce matin même, dans le cadre d'un rappel au règlement, par ma collègue Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale,

Monsieur le président, je n'envisageais pas le moins du monde de prendre la parole, mais je veux simplement dire qu'hier j'ai posé une question d'actualité au Gouvernement sur le fait que, face aux régimes autoritaires, les démocraties paraissaient bien faibles.

pour que notre pays exprime sa position en lien avec nos responsabilités européennes et notre engagement dans une alliance défensive, je considère qu'il est préférable

pays de l'Union européenne. Elle sera l'occasion, cher président Karoutchi, de réaffirmer un certain nombre de principes de manière forte.

Monsieur le Premier président, madame la rapporteure générale, même dans ces circonstances, c'est avec plaisir et un grand intérêt que nous vous accueillons ce matin à l'occasion du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. Au nom du Sénat tout entier, je vous remercie de votre présence. Cet exercice constitue un moment d'échange privilégié et attendu. Comme vous le savez, le Sénat attache une grande importance à la mission d'assistance du Parlement au contrôle du Gouvernement, que notre Constitution confie à la Cour des comptes. Nous avons d'ailleurs pu échanger, monsieur le Premier président, madame la rapporteure générale, sur les conditions qui nous permettront de conforter encore cette mission. Pour la troisième année consécutive, comme nous y autorise la loi organique relative aux lois de finances, le dépôt de votre rapport, monsieur le Premier président, va donner lieu à un débat au cours duquel tous les groupes politiques constituant notre assemblée pourront s'exprimer. J'insiste sur ce point car c'est bien ainsi que notre contrôle démocratique doit s'exercer, dans le respect du pluralisme Cette année, monsieur le Premier président, votre rapport est consacré à la gestion de la crise sanitaire et aux actions mises en oeuvre pour lutter contre ses conséquences économiques et sociales. le dites vous-même, à un moment charnière pour nos finances publiques et notre modèle de croissance économique. Après le très fort recul de 2020, notre économie a rebondi en 2021 et a retrouvé à la fin de l'année dernière son niveau d'avant-crise. Il nous faut maintenant reprendre un chemin de croissance dynamique.

Cette situation exige, dites-vous, des efforts importants de redressement afin d'assurer la soutenabilité de nos finances publiques. a montré la grande réactivité et l'extraordinaire capacité de mobilisation de nos services publics ainsi que d'un grand nombre de secteurs d'activité, mais elle a aussi révélé des vulnérabilités et des risques de dépendance forte vis-à-vis de l'extérieur

Enfin, elle a mis en lumière certaines faiblesses structurelles de notre modèle socioéconomique.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission des affaires sociales,

l'unité s'impose et elle est aussi celle des institutions. Or la Cour des comptes est une institution de la République, qui, vous le savez, contrôle les ministères régaliens, le ministère de l'intérieur, le ministère de la défense et celui des affaires étrangères. nous nous sentons pleinement impliqués dans ce moment. Je vous remercie, monsieur le président, des mots de bienvenue et de l'accueil que vous avez réservé à la Cour, lequel traduit la qualité des liens qui unissent nos deux institutions-

accompli pendant une année charnière dans la lutte contre la pandémie de covid-19 et dans la refonte de notre modèle socioéconomique. Il se structure autour de dix-neuf chapitres thématiques, précédés par un chapitre introductif relatif aux finances publiques. Il s'agit non pas seulement d'analyser nos comportements dans l'urgence, mais d'apprécier

Si cette action était indispensable pour préserver l'activité et pour nourrir la croissance à venir, elle pèsera durablement sur le déficit et la dette publics. Le nécessaire redressement des finances publiques passera également par des efforts importants importants de maîtrise de nos dépenses. Le chapitre introductif du rapport public annuel montre que, si l'année 2021 a été celle d'un très fort rebond de l'activité économique, cette reprise s'accompagne d'un déficit public élevé et structurel. Le déficit public se maintient à 8,2 points de PIB, ramené à 7 points selon les dernières déclarations du Gouvernement ; il serait encore de quelque 5 points en 2022. Ce qui est inquiétant pour l'année 2022, c'est la dimension structurelle du déficit.

Vous l'aurez compris, pour atteindre de tels niveaux de déficit et d'endettement publics, les dépenses publiques françaises ont considérablement augmenté, au-delà même des mesures temporaires, et ont atteint un niveau nettement nettement supérieur à celui d'avant la crise. Les dépenses publiques représenteraient 59,8 % du PIB en 2021 et 55,7 % en 2022 ; elles seraient ainsi supérieures de près de 2 points de PIB à leur niveau de 2019, qui était déjà important. Observons d'ailleurs que nous vivons depuis

qui expliqueraient à hauteur de 2 points de PIB la hausse des dépenses publiques entre 2019 et 2022, c'est bel et bien la mise en place de nouvelles dépenses pérennes qui vient dégrader le solde structurel. S'agissant des recettes, nous soulignons dans le rapport public annuel (RPA) que leur hausse, portée par le rebond de l'activité en 2021, a été freinée par d'importantes baisses d'impôts. En 2021 et 2022, les prélèvements obligatoires augmenteraient respectivement de 5,1 % et de 4,6 %, soit moins que l'activité économique. Le taux de prélèvements obligatoires baisserait donc d'un peu plus de 1 point ces deux années, passant de 44,5 % en 2020 à 43,8 % en 2021 et à 43,4 % du PIB en 2022. L'état des lieux que je dresse devant vous très rapidement doit être pris au sérieux, d'autant que

Un tel objectif ne peut être atteint qu'en menant une politique budgétaire ciblée visant à redresser la trajectoire des finances publiques. Quelles pistes proposons-nous face à ce défi ?

ont été globalement réactifs. Ils ont fait preuve d'une très grande capacité d'adaptation, et même d'innovation, pour protéger la population, pour assurer la continuité du service public et pour préserver le tissu économique. Dans ce rapport, nous leur tirons un coup de chapeau,

Malgré les contraintes initiales qui étaient les leurs et l'intensité de l'activité à laquelle ils étaient confrontés, les acteurs publics ont su se mobiliser rapidement. Je vais vous en donner en donner quelques exemples. Le chapitre relatif à la direction générale des finances publiques (DGFiP) et à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) illustre parfaitement la mobilisation du personnel administratif, le développement des méthodes de travail à distance et la numérisation des procédures.

seuls 27 % des agents de la DGDDI, hors branche surveillance, et 17 % des agents de la DGFiP étaient équipés d'ordinateurs portables en mars 2020.

Comme cela a été fait partout en Europe, l'administration pénitentiaire a accéléré les sorties de détenus condamnés à des peines légères ou présentant les meilleures chances de réinsertion. Nous émettons toutefois une réserve importante concernant la politique vaccinale des détenus et du personnel pénitentiaire, qui n'ont pas été considérés comme prioritaires- à tort, à notre avis. En outre, je voudrais souligner le rôle clé joué par l'État, qui a choisi d'apporter un soutien massif aux secteurs les plus fortement touchés par la crise sanitaire et à l'activité économique du pays.

des PGE. Ce succès a été favorisé par la coopération étroite entre l'administration, les acteurs financiers et Bpifrance. En 2020, les PGE ont largement dominé les autres crédits publics et privés, représentant alors 120,8 milliards d'euros d'encours. L'État a également fait le choix d'intervenir directement dans des secteurs spécifiques, à l'instar du monde sportif. Face à la chute dramatique du chiffre d'affaires du secteur- quelque 20 milliards d'euros en 2020 -, l'État a mis en place des aides importantes en faveur du sport. À l'image de la crise elle-même, il a fallu prendre des mesures fiscales exceptionnelles. Nous montrons, dans un chapitre entièrement dédié à ces mesures, comment l'administration fiscale française a pris les décisions adéquates pour soutenir la trésorerie des entreprises. l'État a été particulièrement présent pour maintenir la bonne gestion des biens de première nécessité, comme l'électricité et les transports collectifs, qui ont été lourdement frappés par la crise. Le maintien de l'alimentation en électricité est un bel exemple de coopération et de coordination entre les acteurs publics et privés du secteur électrique.

Île-de-France Mobilités et les opérateurs ont subi, de ce fait, de très grosses pertes financières liées à la contraction des recettes tarifaires, mais l'État a accepté de les compenser massivement. Il me semble important de rappeler que c'est cette présence positive de l'État

de signes de dégradation. Dans le même esprit, le chapitre relatif aux mesures européennes en faveur de l'emploi fait ressortir des lacunes dans le pilotage du ministère chargé du travail. La France se singularise par une dispersion des financements vers une multitude d'actions et de porteurs de projets, ce qui complique la gestion et l'audit des fonds correspondants. La culture de la maîtrise des risques doit être renforcée dans notre pays. Plus globalement, il ressort de nos travaux que le manque de calibrage des dispositifs pourrait provenir d'une insuffisante connaissance de leurs bénéficiaires potentiels. Un chapitre très important sur les dispositifs de soutien à la vie étudiante déplore la prise en charge tardive de la communauté étudiante lors de la crise. Ce retard reflète l'éloignement et le manque de données et d'informations sur la population des étudiants. Les dispositifs retenus ont été essentiellement dirigés vers des publics connus, à savoir les boursiers.

je tiens à évoquer en priorité les travaux réalisés par les chambres régionales et territoriales des comptes. Ceux-ci mettent en lumière l'articulation parfois difficile des interventions des acteurs publics nationaux et locaux. Le chapitre dédié aux interventions économiques des collectivités locales d'Occitanie

morte. Chaque niveau de collectivité a développé son propre mécanisme de soutien, parfois au prix d'une stratégie de contournement des règles définissant ses compétences. Le chapitre relatif au contrôle des délégations de service public dans les Hauts-de-France souligne, quant à lui, que, faute d'une stratégie claire face aux impératifs de continuité et d'adaptation du service public, les autorités délégantes ont trop souvent accédé sans réelle discussion aux demandes des entreprises délégataires, malgré la chute des activités déléguées et la baisse de la qualité de service aux usagers. Enfin, nous déplorons que les aides accordées n'aient généralement pas été assorties de précautions suffisantes pour éviter des effets d'aubaine ... Ah ! ... et limiter les risques de fraude. Bravo ! Le suivi des mesures fiscales exceptionnelles, dont j'ai déjà souligné toute la pertinence, était difficile en raison des rigidités liées au système d'information de l'administration fiscale. Une attention similaire doit être prêtée au suivi des

De manière plus sectorielle, nous identifions des limites similaires pour les aides de l'État en faveur du mouvement sportif. Les moyens dédiés aux contrôles ont été quasi inexistants et le déploiement des aides s'est fait dans une grande confusion entre les mesures d'urgence et les mesures de relance.

adopter. Le troisième et dernier enseignement que je veux tirer de ce RPA 2022 est que les faiblesses structurelles de notre système productif et de notre modèle social et de transition écologique ont été accentuées pendant la crise sanitaire. La pandémie a d'abord rappelé que nous étions individuellement et collectivement vulnérables. Notre première vulnérabilité réside évidemment dans la production de produits de santé. La hausse brutale de la demande, en particulier concernant les médicaments ou les masques de protection sanitaire, a mis à mal le fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement. Le chapitre du RPA relatif à l'approvisionnement en produits de santé démontre que les pénuries auxquelles nous avons été confrontés exposent au grand jour notre dépendance- désormais bien documentée -à l'égard de certains produits importés.

J'ai une pensée particulière pour les 600 000 résidents des Ehpad, qui figurent parmi les personnes ayant le plus souffert de la crise. Entre mars 2020 et mars 2021, la pandémie a provoqué près de 34 000 décès

je souhaite évoquer un thème d'une très grande importance, celui de la transition écologique. Nous avons choisi d'illustrer les répercussions du changement climatique au travers de la situation des stations de moyenne montagne des Pyrénées-Atlantiques.

: lorsque l'on aborde la crise sanitaire et les préoccupations des Françaises et des Français, il n'y a pas de petit sujet. Le rapport dresse un tableau objectif de la France en sortie de crise, avec des forces et des faiblesses, des défis à relever ainsi que des atouts et des lacunes. Je veux être optimiste, avec l'optimisme de la volonté, mais aussi celui de la rationalité.

Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, la remise du rapport public annuel est un moment important, car elle symbolise l'assistance que la Cour des comptes apporte au Parlement, laquelle dépasse largement le cadre de la présentation d'aujourd'hui. Chaque année, la commission des finances mène des contrôles budgétaires, dont certains s'appuient sur les résultats d'enquêtes qu'elle demande à la Cour en application de l'article L. 58-2 de la loi Hier encore, notre commission a entendu les magistrats de la Cour venus lui présenter son enquête sur les mesures de soutien à l'industrie aéronautique. La qualité de cette enquête, qui incluait des cahiers territoriaux, a été unanimement saluée. Nous entendrons de nouveau la Cour au début du mois de mars sur l'élaboration, le pilotage et la mise en oeuvre des crédits du plan de relance, puis avant la suspension estivale sur les dépenses de l'État pour l'outre-mer. outre, nous attendons avec intérêt la remise, au mois de septembre prochain, d'une enquête sur les scénarios de financement des collectivités territoriales, en vue de l'examen à l'automne d'un projet de loi de programmation de nos finances publiques, un événement qui n'a pas eu lieu depuis cinq ans. J'en viens maintenant au contenu du rapport public annuel. Le RPA dépeint tout d'abord une situation de nos finances publiques que nous connaissons bien, pour l'avoir suivie au cours de nos travaux sur les lois de finances initiale et rectificatives.

Les dépenses de crise, comme l'activité partielle, le fonds de solidarité ou encore les mesures de relance, dont le montant s'est élevé à 70 milliards d'euros en 2020 et 90 milliards d'euros en 2021, étaient évidemment nécessaires.

pour sécuriser la soutenabilité de notre dette. Sans cette érosion des recettes publiques, notre dette aurait été inférieure d'environ 6 points de PIB par rapport à son niveau attendu en 2022, ce qui représente près de 160 milliards d'euros. À ce jour, je crois pouvoir dire que les effets prétendument positifs de ces réformes fiscales, notamment celles de l'impôt sur la fortune, du prélèvement forfaitaire unique, comme celle des impôts de production, sont pour le moins peu documentés. Il me paraît donc important de faire preuve de mesure dans la manière dont nous abordons les années qui s'annoncent sur le plan de nos finances publiques. Je remarque le retour d'une musique bien connue et qui nous appelle à une maîtrise « renforcée », « stricte », « sans faiblesse », « urgente » de nos dépenses publiques. qu'ici ou là certains préconisent en même temps une nouvelle baisse des prélèvements en la gageant par des réformes « structurelles », dont on peine en réalité à saisir les contours. Certes, je suis comme vous attentif aux risques pesant à terme sur notre soutenabilité budgétaire. Ceux-ci pourront d'ailleurs être réexaminés prochainement compte tenu de l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt. notre principal objectif doit être d'abord de soutenir notre croissance, le pouvoir d'achat des ménages et l'investissement. Or, comme nous l'avons vu dans le passé, un ralentissement ou une baisse brutale des dépenses aurait des effets très négatifs sur l'activité économique : ces éléments doivent être pris en compte, notamment au niveau européen. Comme toujours, le RPA comprend des insertions thématiques, qui font souvent écho aux observations formulées par nos rapporteurs spéciaux. La Cour analyse ainsi les dispositifs déployés par l'État pour accompagner les étudiants. Comme le relevait notre collègue Vanina Paoli-Gagin dans son rapport budgétaire,

Dans ce contexte, les mesures d'urgence mises en place ont souffert d'un ciblage inadéquat ; à titre d'exemple, le repas à 1 euro, créé en septembre 2020 au profit des seuls étudiants boursiers, n'a été généralisé de janvier 2021 à l'ensemble des étudiants. Ce constat invite à développer une connaissance plus fine de cette population, afin de créer des dispositifs mieux adaptés à ses besoins. La Cour dresse aussi un bilan de l'efficacité du plan « 1 jeune, 1 solution ». Ce plan a contribué à modifier la structure de l'emploi : aux contrats très courts et d'intérim

entre les différents acteurs du service public de l'emploi. Elle rejoint ainsi pleinement les constats formulés à plusieurs reprises tant par le rapporteur spécial des crédits de la mission « Plan de relance », Jean-François Husson, que par les rapporteurs spéciaux de la mission « Travail et emploi », Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian. Comme ces derniers l'avaient d'ailleurs souligné, le nouveau contrat d'engagement jeune, qui remplace la garantie jeunes, contribue à rationaliser cette politique, mais sa mise en oeuvre, introduite par voie d'amendement sans étude d'impact ni d'ailleurs de débat parlementaire, reste entourée de fortes incertitudes. S'agissant des grands aéroports français, la Cour pointe les limites d'un modèle économique qui reposait sur la perspective d'une forte croissance du trafic. Elle souscrit ainsi au constat et aux pistes formulées par notre collègue Vincent Capo-Canellas ... Excellent ! ... dans son dernier rapport budgétaire, en relevant l'impasse du modèle de financement actuel des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Ce système, qui repose sur une taxe affectée dont le rendement a été fortement minoré par la crise, menace l'équilibre financier des aéroports. L'État leur a accordé des avances remboursables, qui ne font, selon nous, que repousser le problème. Vincent Capo-Canellas avait à cet égard pris une position plus explicite en considérant que les conséquences de la crise sur le déficit de financement de ces missions régaliennes devaient être assumées par l'État sous forme de subventions.

Le rapport souligne que leur coût final est incertain et dépendra de l'évolution de la situation financière des entreprises. Il insiste sur la nécessité de porter une attention particulière aux risques d'optimisation des PGE. Alors que la

de soutien aux entreprises sont examinés dans un titre spécifique du RPA, qui revient à la fois sur les mesures de report, de baisse exceptionnelle et les aménagements dits de « bienveillance Je souscris au constat de la Cour d'un suivi parfois complexe de ces dispositifs. Alors que les reports d'échéances fiscales ont fait l'objet d'une conditionnalité limitée- absence de versements de dividendes, de rachats d'actions ou encore de siège ou de filiale dans un État ou un territoire non coopératif -j'insiste sur la nécessité

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, comme chaque année, notre commission a pris connaissance avec grand intérêt du rapport public annuel que la Cour des comptes a publié le 16 février Cette publication intervient après deux années de pandémie et à la veille de l'élection présidentielle et des élections législatives. Dans un tel contexte, les constats et les préconisations de la Cour prennent un relief particulier. Tout d'abord, s'agissant des comptes publics, la Cour souligne que, malgré le fort rebond de l'économie française en 2021, notre pays, entré dans la crise avec l'un des plus forts déficits de l'Union européenne, n'en sortira pas en meilleure posture. J'observe que ce constat vaut également pour les comptes sociaux. En effet, les comptes de la sécurité sociale n'étaient pas revenus à l'équilibre lorsque la pandémie a éclaté et les perspectives sont inquiétantes. J'ai bien noté qu'en s'exprimant aux côtés d'Olivier Dussopt devant les commissions des affaires sociales et des finances de l'Assemblée nationale, le 26 janvier dernier, Olivier Véran a estimé que les déficits cumulés de la sécurité sociale pourraient dépasser 300 milliards d'euros durant la décennie 2020-2030, soit une moyenne de déficit de 30 milliards d'euros par an et un cumul de déficit qui dépasserait de quelque 200 milliards de la dette sociale (Cades) au titre des déficits postérieurs à 2019- excusez du peu ! Dans ces conditions, on comprend mieux le refus obstiné du Gouvernement d'intégrer une règle d'or dans le cadre organique des futures lois de financement de la sécurité sociale, comme l'a proposé le Sénat. Nous aurons l'occasion d'en reparler en détail avec le ministre délégué aux comptes publics, que nous entendrons le 15 mars prochain. En plus de ces observations macroéconomiques, la Cour des comptes a conduit diverses études thématiques, dont plusieurs fournissent des éléments précieux à la commission des affaires sociales. le Premier président, vous avez insisté à juste titre sur les tensions importantes observées ces dernières années sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Nous avons tous en tête le manque de masques et la grande peur du printemps 2020 sur le risque de pénurie de curares, d'hypnotiques injectables et même de paracétamol. le Sénat avait mis en garde contre l'augmentation des ruptures de stock, touchant aussi bien les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur que ceux d'usage quotidien. Constatant un risque de déstabilisation de notre système de soins,

aux décisions d'urgence prises pendant la crise ou encore à la modification des conditions de détermination des prix en 2021 pour inciter au maintien de la production des médicaments anciens.

La Cour préconise de donner un rôle plus actif à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans la définition des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et, pour les plus indispensables d'entre eux, appelle à une action plus énergique pour prévenir les tensions d'approvisionnement. Le Sénat souscrit à ces recommandations. Mais celles-ci doivent impérativement s'accompagner d'un soutien actif à la localisation en France et en Europe : tel était le sens des amendements de notre commission déposés sur Le rapport public annuel consacre également des développements à la question des personnes âgées hébergées dans les Ehpad, car il vous a paru utile de rendre compte des conséquences de la crise sur ces établissements. Il est impossible de ne pas s'arrêter quelques instants sur ce sujet, qui trouve un écho particulier à la suite de la publication de l'ouvrage du journaliste Victor Castanet et de l'émotion légitime que celui-ci a suscitée. Notre commission a d'ailleurs décidé de créer une mission d'information dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête afin d'analyser les procédures et la politique de contrôle déployées dans ce secteur. Hier, elle a reçu hier les conclusions d'une enquête demandée à la sixième chambre de la Cour relative à la médicalisation des établissements. Le rapport pointe le lourd bilan humain provoqué par la pandémie de covid-19 sur les personnes âgées ; je m'associe à la douleur des familles. Ce bilan n'est pas imputable à la seule vulnérabilité particulière des personnes âgées dépendantes : les taux d'encadrement dans la prise en charge de ces personnes ont aussi des effets majeurs. La crise est le révélateur d'une problématique qui n'est malheureusement pas nouvelle. Nous souscrivons à cette analyse, que nous nous attachons à approfondir par nos travaux réguliers sur la politique de l'autonomie, en collaboration avec la Cour, à qui nous avons demandé dans les derniers mois deux enquêtes sur ces sujets. Quelles sont les faiblesses structurelles les plus importantes ? Votre constat est clair : les Ehpad les plus touchés sont ceux dont la proportion de personnel paramédical, d'infirmiers ou de médecins coordonnateurs était la plus basse. En approfondissant votre analyse, vous observez également que les Ehpad privés commerciaux, pour lesquels le taux d'encadrement des résidents est moins élevé, ont été significativement plus touchés que les autres structures lors de la deuxième vague de l'épidémie. Il ne s'agit évidemment pas de jeter l'opprobre sur un secteur, mais il convient de souligner la convergence des analyses sur le fait que la qualité des prises en charge dans les Ehpad est bousculée par les fortes tensions sur les personnels, en période de pandémie plus encore qu'en période normale. des efforts ont été faits : le taux d'encadrement dans les Ehpad s'est amélioré depuis dix ans et le Ségur de la santé a contribué à une amélioration des conditions salariales, mais, pour reprendre l'expression utilisée par la Cour, qui se caractérise par une insuffisance du taux d'encadrement, une mauvaise organisation des cycles de travail, un absentéisme élevé et un manque de formation, suscite de réels problèmes de qualité des prises en charge. Nous serons attentifs à ce que des solutions nouvelles et complémentaires soient mises en oeuvre pour réduire ces tensions. En matière d'emploi des jeunes, vous avez examiné les conditions de déploiement, les premiers résultats ainsi que les coûts du plan « 1 jeune, 1 solution ».

en passant par la réactivation de contrats aidés qui avaient pratiquement disparu ou qui ne ciblaient plus prioritairement les jeunes. Initialement doté de 6,5 milliards d'euros, » aura coûté, selon votre rapport, près de 10 milliards d'euros pour les années 2020 et 2021, dont près de 6 milliards d'euros pour les seules aides à l'embauche en alternance. Il faut reconnaître la mobilisation du ministère du travail, ainsi que la coordination entre les acteurs dans la mise en oeuvre de ce plan. La situation de l'emploi des jeunes a été préservée, puisque le taux de chômage est de 20 % chez les 15-24 ans au troisième trimestre 2021, en baisse de 1,2 point par rapport à son niveau d'avant-crise. La part des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation- les NEET -a quant à elle diminué de 0,8 point, à 11,6 %. Toutefois, votre rapport est très réservé quant à l'impact direct du plan « 1 jeune, 1 solution » sur cette situation favorable. En particulier, l'effet net sur l'emploi des aides à l'embauche a vraisemblablement été faible, même si celles-ci ont permis une amélioration de la qualité des emplois. Vos observations sur les dispositifs d'accompagnement intensif, notamment la garantie jeunes, ont retenu toute notre attention. Il semble qu'un changement d'échelle expose ces dispositifs à des risques de perte de substance et d'efficacité. Ainsi, Ainsi, les résultats en termes d'insertion dans l'emploi de la garantie jeunes, déjà fragiles en temps normal, se sont dégradés pendant la crise avec moins de 20 % d'entrées dans l'emploi. La proportion de jeunes ayant bénéficié d'une période d'immersion dans le monde du travail au cours de leur parcours a été divisée par deux. Ce constat doit nous inciter à la vigilance, alors que le nouveau contrat d'engagement jeune, qui cible 400 000 jeunes contre 100 000 contrats en vitesse de croisière pour la garantie jeunes, doit être mis en place dans quelques jours : il n'est pas souhaitable que ces dispositifs soient dilués dans une sorte de « RSA jeune ». La remobilisation des contrats aidés s'est révélée laborieuse, notamment sous la forme des parcours emploi compétences (PEC) jeunes dans le secteur non marchand. Il convient de s'interroger sur la pertinence de ces outils en tant que réponse conjoncturelle à la crise. À cet égard, nous soutenons votre recommandation d'évaluer leur valeur ajoutée en termes d'insertion

le rapport public annuel de la Cour des Comptes tire un bilan des enseignements de la crise et de ses conséquences budgétaires, financières, économiques et sociales. J'en partage les constats,

Le plan de relance a irrigué l'économie, la maintenant à flot avec une efficacité hors norme dans certains secteurs, comme celui de l'hôtellerie-restauration. Malgré des fermetures prolongées,

n'en avoir dépensé qu'une faible part. Le Gouvernement devrait être en mesure de tracer cet argent pour éviter qu'il ne se perde et s'assurer qu'il soit investi à bon escient pour développer notre économie. économie. Monsieur le Premier président, le rapport de la Cour s'intéresse aux collectivités territoriales d'Occitanie. Il souligne le manque d'efficacité de l'intervention des régions et des départements pour soutenir les entreprises du fait de l'existence préalable d'une aide nationale. De plus, compte tenu de la faiblesse des taux de remboursement pour la commande publique, ce levier n'a pas apporté de grands bénéfices aux entreprises. Ainsi, selon le rapport, la multiplication des dispositifs a été « peu propice à l'efficience » et « peu sécurisée au plan juridique ». Mais il ne faut pas oublier le contexte.

À mon avis, la solution est non pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux. Un euro dépensé doit être un euro utile. À l'image d'une fuite au niveau d'une canalisation d'eau, une part importante de la dépense publique se perd dans des frais généraux qui ne contribuent pas à la réalisation de missions de service public. Il faudrait fixer une règle d'or à nos administrations, en limitant la part de ces frais généraux. Dépenser mieux signifie que l'on doit utiliser l'argent public pour atteindre le but recherché. Le budget du ministère de la santé doit servir pour soigner, et non pour financer une myriade de structures administratives. Il en est de même pour l'éducation nationale. Prenons l'exemple de l'école de ma commune où travaillent trois enseignants. Sa directrice est détachée à mi-temps pour effectuer des tâches administratives. Celle-ci me confiait il y a peu que, face aux flux d'enquêtes, de questionnaires et autres paperasseries, elle n'y parvenait pas

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, comme chaque année, le rapport public annuel de la Cour présente des éléments sectoriels très intéressants. Ma collègue Isabelle Briquet reviendra au nom

en coûte » mis en place pour répondre à cette crise, n'est pas souhaitable. C'est l'un des enseignements de la sortie en partie manquée de la crise de 2008. Je note aussi la critique de la Cour sur la qualité des prévisions budgétaires du Gouvernement, qui pose question.

moins mauvais que prévu, est présenté comme une bonne nouvelle, est trompeur vis-à-vis des citoyens comme du Parlement. Nous l'avions d'ailleurs dit lors de la discussion budgétaire.

l'explosion des profits de certaines grandes entreprises, la hausse de la distribution des dividendes et l'importance des aides à la production sans aucune conditionnalité. Il faut donc réfléchir- les socialistes n'ont cessé de le dire -non seulement aux dépenses, mais aussi aux recettes, en particulier à l'utilité de chacune des niches fiscales, qui grèvent les recettes de l'État. Un levier a été identifié par le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport sorti au début du mois, celui d'une réforme en profondeur du crédit d'impôt recherche.

la question des droits de succession revient sur le devant de la scène, c'est-à-dire celle de la reproduction des inégalités de patrimoine. Il y a tant de progrès à faire en ce domaine, sans pour autant entraver la croissance. Pendant cinq ans, le Gouvernement s'est entêté à mettre en oeuvre une politique de l'offre,

Mais dès avant la crise, les bases étaient très dégradées, car le « ruissellement » était resté un mythe et l'État avait été appauvri par une politique fiscale injuste. Il est donc nécessaire d'en finir avec le « en même temps » budgétaire, qui creuse le déficit et reporte les dépenses sur les générations futures. Il est temps de mettre enfin de la cohérence dans la gestion des finances publiques, de faire des choix politiques courageux et qui ne se limitent pas aux dépenses. Tel est l'enjeu qui est aujourd'hui devant nous.

depuis 190 ans, la Cour des comptes remet chaque année son rapport public annuel. Celui-ci constitue désormais un rendez-vous incontournable de notre vie démocratique et une vigie financière pour l'État et ses administrations. Ce n'est pas un hasard si l'avis de la Cour est respecté de tous ; ses rapports n'hésitent pas à pointer les insuffisances des administrations publiques, afin d'orienter l'État et les gouvernements qui se succèdent, tous autant qu'ils sont, dans le but d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. L'an dernier, à cette même tribune, je rappelais les deux principaux axes du rapport 2021, qui, soulignait que la crise avait révélé les fragilités structurelles de l'État et de ses opérateurs, et qui, d'autre part, saluait la réactivité inédite de nombreuses administrations et organismes publics ayant su s'adapter avec une remarquable énergie. Cette année, le rapport que remet la Cour s'inscrit une fois encore dans cet esprit. Les constats sans appel qu'elle présente nous invitent à la vigilance. Comme l'a rappelé le Premier président devant l'Assemblée nationale, « il ne s'agit pas seulement d'évaluer notre action dans l'urgence, mais d'apprécier notre résilience et notre capacité à remédier aux faiblesses structurelles que la crise a révélées ou accentuées ». C'est précisément ce point que je souhaite développer devant vous. Je commencerai par l'un des principaux enseignements de ce rapport. Nous faisons face à un problème structurel : chaque crise crée un effet de cliquet sur les dépenses publiques. À l'issue de la crise, les dépenses, y compris structurelles, se retrouvent toujours plus élevées

des marges de manoeuvre budgétaires en période de croissance, ce qui nous permettra d'apporter une réponse d'ampleur en cas de crise sans menacer pour autant l'équilibre à moyen et long terme de nos finances publiques.

Mes chers collègues, en réalité, nous devons agir sur chacun des secteurs de l'action publique, à l'image de la réflexion de la Cour, qui, au travers de dix-neuf chapitres, aborde différents sujets sectoriels, soit parce que les enjeux sont particulièrement décisifs, soit parce qu'ils illustrent avec justesse les problèmes structurels dont nous parlions. Bien souvent, ces problèmes ne sont pas récents. Quand ils le sont, ils trouvent leur origine dans des décennies d'incurie et de négligence de la part des pouvoirs publics et des gouvernements successifs. protéger nos concitoyens de leurs conséquences, et ce n'était pas au plus fort de la crise que nous pouvions les résoudre. Mais, aujourd'hui, il est essentiel de tirer les enseignements de cette pandémie pour y répondre durablement dans les mois et années à venir. Parmi ces sujets, j'en évoquerai deux qui me tiennent particulièrement à coeur : les aides au secteur sportif et le soutien apporté aux stations de moyenne montagne. La Cour a souligné le « volontarisme de l'État » et des collectivités durant la crise en faveur du monde sportif. Néanmoins, ce secteur souffre de longue date de son éclatement et de la multiplication des interlocuteurs institutionnels, qui qui rendent difficile une réponse claire et uniforme. C'est un problème que je connais également bien en tant que rapporteur spécial des crédits de la mission « Culture ». Dans ce domaine comme dans celui du sport, il nous faudra élaborer les outils permettant de suivre au plus près l'action de l'État et des collectivités, ce afin de doter les pouvoirs publics de véritables instruments de pilotage des aides et de rendre plus lisibles et plus efficaces la multitude de dispositifs mis en place, qu'il s'agisse d'apporter un soutien structurel ou de répondre aux crises qui pourraient survenir. Nous touchons là à un enjeu de contrôle et d'évaluation des politiques publiques et sommes au coeur de notre rôle de parlementaires. des stations de moyenne montagne, là encore le problème n'est pas nouveau et la crise a agi comme un révélateur de leur fragilité grandissante. Je l'ai constaté dans mon département, en Isère, au plus fort de la crise. Il est indispensable que que nous travaillions à réinventer leur modèle économique et que nous accompagnions leur transformation pour les aider à retrouver leur santé financière. C'est toute l'ambition du plan Avenir montagnes, que je suis avec attention depuis son lancement. Enfin, je ne peux évidemment pas faire l'impasse sur la gestion de la crise dans les Ehpad. Faiblesse du taux d'encadrement, faiblesse de la médicalisation, vétusté des équipements, les difficultés structurelles sont nombreuses. L'effort de l'État est pourtant considérable et en nette augmentation

trop longtemps éloigné du contrôle de l'État. Le récent scandale qui a éclaté en est la triste preuve. Tels sont les défis qui nous attendent et qui devront occuper nos débats au cours des semaines qui viennent. Il s'agit d'enjeux fondamentaux pour notre démocratie, pour la continuité de l'action de l'État et pour les générations à venir.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, l'actualité a ceci de singulier qu'elle peut changer du tout au tout en quelques jours. Aujourd'hui, nos regards sont, à raison, rivés vers l'Est, où la Russie ravive les peurs d'un conflit mondial, mais aussi vers le Sud, où la situation malienne nous fait craindre l'émergence d'une nouvelle base djihadiste. Quand la situation internationale cesse de nous occuper, nous en revenons à nos affaires nationales. Alors, les prochaines échéances électorales saturent tout l'espace médiatique. Nous en arrivons à oublier qu'une pandémie bouleverse le monde depuis deux ans. Pourtant, s'il y a bien un domaine où nous ne sommes pas près d'oublier la crise sanitaire, ce sont nos finances publiques. Le rapport public annuel de la Cour des comptes constitue en cela une douloureuse piqûre de rappel. Tous les principaux indicateurs prouvent que nos finances publiques ont été lourdement éprouvées par la crise. Notre déficit demeure extrêmement élevé, autour de 130 milliards d'euros en 2022,

au-dessus du niveau de 2019. Notre pays demeure le champion des prélèvements obligatoires et de la dépense publique, même si les taux sont, en l'occurrence, déjà revenus au niveau d'avant-crise. Une simple analyse de ces indicateurs nous rappelle que la France mettra des années, si ce n'est des décennies, pour effacer de ses comptes publics les séquelles de la pandémie. Nous paierons longtemps les mesures d'urgence. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler ces éléments structurants, non pas pour accabler le Gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire, mais parce que le désendettement de l'État doit devenir une priorité politique pour les prochaines années. Il y va de notre souveraineté nationale. Le creusement du déficit et de la dette publique est dû à une hausse très forte des dépenses et à une baisse très forte aussi des recettes. Or c'est le même phénomène qui s'applique à plusieurs échelons. Je souhaite évoquer ici le cas des grands aéroports, qui fait l'objet d'un chapitre à part entière du rapport public annuel de la Cour des comptes. Là encore, l'effondrement des recettes et l'augmentation des dépenses ont fragilisé les structures. Avec la crise, le trafic aérien a connu un coup d'arrêt brutal. Certains scénarios indiquent qu'il faudra attendre 2024 en Europe pour que le trafic aérien retrouve son niveau d'avant-crise. En conséquence, les recettes des aéroports, qui dépendent directement du trafic, se sont elles aussi effondrées et, avec elles, les marges d'exploitation. Le soutien de l'État a été total, mais les aéroports ont été contraints à de grands plans d'économie pour assainir leurs finances. Plus fondamentalement, c'est tout un modèle qui est remis en question. Le rapport public annuel a mis en évidence les limites du financement par la taxe d'aéroport des missions de sécurité et de sûreté. Il faudra repenser l'avenir des aéroports en France après la levée progressive des restrictions sanitaires. Cette situation est d'autant plus grave que la santé financière des aéroports révèle le dynamisme de nombreux territoires. C'est particulièrement le cas chez moi, dans l'île de La Réunion, où l'aéroport Roland-Garros est un poumon économique. Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement sur les deux recommandations formulées par la Cour des comptes à ce sujet. Pour les élus de La Réunion, il s'agit non pas seulement de savoir si les comptes de notre aéroport seront équilibrés, mais bien de savoir si notre île pourra retisser plus fortement les liens humains, commerciaux et économiques

avec la bonne gestion financière d'avant-crise. C'est l'une des conditions du redressement économique de la France. Notre défi sera de nous assurer que cette gestion financière ne se fera pas au détriment de la croissance économique. La parole est

Vincent Segouin. Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, je tiens avant tout à vous remercier pour la rédaction de ce rapport et la qualité de votre travail, qui participe à la transparence de la vie publique et qui nous éclaire. Par votre rapport, vous nous alertez sur le fait que, si l'activité économique de la France a dépassé son niveau d'avant-crise, notre pays connaît néanmoins un déficit structurel sans précédent, équivalent à 5 % de notre PIB, et une dette publique à hauteur de 113,5 % de notre PIB. Ces chiffres sont la conséquence des baisses des prélèvements obligatoires et de la mise en oeuvre de nouvelles dépenses publiques pérennes en 2021 et 2022. Au sein de la zone euro, la France fait dorénavant partie des mauvais élèves qui ne respectent pas la règle d'or, à l'inverse de pays comme l'Allemagne,

La France doit impérativement cesser la politique mortifère de la désindustrialisation et faire du travail et du mérite une priorité. Mardi dernier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, nous a avoué, en commission des finances, que le déficit sans précédent de notre balance commerciale était le point noir, mais qu'il était pour moitié lié à la hausse du coût de l'énergie. Il a de nouveau occulté la baisse de compétitivité des entreprises et la politique énergétique désastreuse menée par le Gouvernement au cours de ce quinquennat. Le nucléaire en est le parfait exemple. Je pense à la fermeture de Fessenheim en début de mandat, qui a marqué la fin du nucléaire en France, puis à cette volte-face à deux mois de l'échéance présidentielle. Pendant que nous achetions de l'énergie carbonée à l'Allemagne, nous n'investissions plus dans la recherche et l'innovation, pourtant garantes de notre efficacité et de notre avenir énergétique. Que de temps perdu ! Que d'argent perdu ! Cette politique à court terme ne sert pas les Français : l'intérêt électoral passe avant, mais à quel prix ? Aujourd'hui, notre balance commerciale est fortement déficitaire déficitaire à cause d'une politique de protection du pouvoir d'achat qui a été menée au détriment du travail et du mérite. Aujourd'hui, 17 % des jeunes ne travaillent pas et n'étudient pas. Le confort des aides sociales leur a fait oublier l'exigence qui veut que, pour avoir de l'argent, il faut produire de la richesse Je m'inquiète pour notre avenir ... Nous n'encourageons plus le mérite et ne reconnaissons plus la valeur du travail. Nos entreprises délocalisent ou se font racheter pour aller produire à bas coût à l'étranger. C'est la conséquence directe du coût de la main-d'oeuvre, des normes, des impôts et des taxes. Augmenter à nouveau ces prélèvements ne ferait qu'amplifier la dégradation de la balance commerciale. Nous continuons à désavantager nos entreprises en produisant trop de normes et en surtransposant, pratiques que ce gouvernement avait pourtant promis de faire cesser.

il a diminué les impôts sur les sociétés, et le montant des prélèvements obligatoires est alors passé de 45 % à 43,5 %. Mais cette diminution n'a de sens au regard de la dette que si les dépenses publiques baissent dans le même temps. Or cela n'a jamais été le cas, bien au contraire

Il est donc nécessaire, comme vous le mentionnez, de réduire les dépenses publiques de 9 milliards d'euros supplémentaires par an. Pour ce faire, il faut réformer, mais ce n'est pas le fort de ce gouvernement- je tiens à le dire. Souvenez-vous de la réforme des retraites, entre autres Je constate que le Gouvernement n'est jamais parvenu à faire des économies dès lors qu'il a été question de prendre le risque de diminuer le confort des Français. Encore une fois, l'exécutif ne pense qu'à court terme et relègue ces mesures impopulaires à ses successeurs. Or la France ne peut plus se le permettre, car la dette que nous avons contractée nous y oblige.

Mais, comme le disait fort justement le président Raynal, la situation serait certainement autre si nous ne nous étions pas privés de recettes fiscales

Alors que l'Insee nous apprend que la France affiche désormais un taux de pauvreté inédit depuis 1979, j'avoue ne pas comprendre les cinq priorités de redressement proposées par la Cour

a réduit les impôts des plus riches, notamment des 10 % les plus riches et, surtout, des 1 % les plus riches, tout en appauvrissant les plus pauvres des Françaises et des Français.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, la Cour des comptes aborde de très nombreux sujets dans son rapport public annuel. Aussi, dans les cinq minutes de temps d'expression qui nous sont alloués, je n'évoquerai qu'un seul sujet, celui de la dette publique. En effet, elle est devenue au fil des années la clé de voûte de l'architecture budgétaire de la France, et gare à celui ou celle qui s'affranchirait des contraintes qu'elle engendre. du 12 avril 2020, au tout début de la pandémie, le Fonds monétaire international (FMI) avait trouvé naturel que les gouvernements adoptent la stratégie du « quoi qu'il en coûte », en précisant toutefois qu'ils devaient bien veiller à conserver les factures. Ce relâchement budgétaire fut une sorte de parenthèse. Aujourd'hui, les financiers nous disent que l'ordre ancien doit retrouver ses droits et la dette, sa fonction, celle qui consiste à discipliner les États dispendieux et les peuples impécunieux. Vous vous souvenez sans doute, mes chers collègues, de la teneur des débats ici même en novembre 2019, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2020. À l'époque, les ministres nous rappelaient que le ratio de la dette sur le PIB en France était de 98,4 %. Nous approchions de la barre fatidique des 100 %. Nous étions au bord de l'apocalypse et, six mois plus tard, pandémie oblige, nous avions atteint les 117 %. En 2004, M. François Bayrou déclarait : « S'il s'agissait d'une entreprise, la France serait au bord du dépôt de bilan. » En 2007, Mme Ségolène Royal déclarait : « La dette publique est devenue insoutenable. » Cette année-là, la dette atteignait 64,6 % du PIB. La dette atteint aujourd'hui environ 115 % du PIB. Toutes les règles ont explosé au cours des deux dernières années : les 3 % de déficit, les 60 % de ratio de la dette ; c'était le monde d'avant ! Ces déclarations catastrophistes et anxiogènes devraient également inquiéter les marchés financiers, ceux qui nous prêtent. Or, il n'en est rien. Avec une telle dette, la France a emprunté très facilement 260 milliards d'euros en 2020, autant en 2021 et la même chose est prévue pour cette année 2022. Vous avez sans doute rencontré

Voyons ce que nous dit le site de l'Agence France Trésor (AFT), qui vend notre dette sur les marchés financiers. Prenons la dernière adjudication en date, celle de lundi dernier, 21 février. Pour les bons du trésor à 3 mois, le taux négatif proposé est de-0,680 %. Pour ceux à 12 mois, il est de-0,585 %. Pour les obligations à terme à 8 ans, nous avons un taux de 0,30 %. Il y a même une obligation à 3 ans qui nous a été proposée à un taux de-0,08 %. Quel étrange paradoxe tout de même, mes chers collègues, de voir ce contraste saisissant entre l'inquiétude orchestrée et l'extrême quiétude des marchés financiers ! C'est à ce titre que j'opposerai, au confort des aides sociales évoqué par notre collègue Vincent Segouin, l'extrême confort des marchés financiers. On peut s'interroger sur la santé mentale des acteurs des marchés. Sont-ils devenus fous ? Sont-ils devenus incompétents ? Ou alors, dans une vision plus humaniste, auraient-ils été soudain touchés par la grâce pour se tourner désormais vers l'action philanthropique et l'amour du prochain ? Permettez-moi de ne retenir aucune de ces trois options. La réponse à cet apparent paradoxe, je crois l'avoir trouvée dans un reportage diffusé sur la radio de service public France Inter, le 20 janvier 2021. La scène se déroule dans les locaux de l'Agence France Trésor à Bercy. Ce jour-là, l'AFT vend 6 milliards d'euros de dette et voici ce que déclare à la journaliste le directeur général de l'époque, M. Anthony Requin : « La France a un très bon crédit auprès des investisseurs, une rente jusqu'à 10 fois supérieure à l'offre, la dette française fait office de valeur refuge, un coffre-fort qu'elle fait payer. « Les gens placent leurs économies pour être sûrs de récupérer leur somme et un coffre-fort, ça se loue. Les investisseurs nous confient leurs liquidités, ils paient le prix de la location de cette sécurité, c'est le taux d'intérêt négatif que vous voyez. Le coffre-fort, c'est la signature de l'État.

à qui fut imposée une purge budgétaire insupportable en 2010, au moment de la crise. À cette époque, son ratio de dette sur PIB était de 147,5 %. Dix ans plus tard, ce ratio est passé à 206,3 %. Le dernier mot reviendra à notre ancien collègue, Jean-Pierre Raffarin. Raffarin. Le 7 juillet 2011 sur RTL, il expliquait : « Au fond, dans le passé, l'élection présidentielle dépendait d'un seul facteur, l'avis des électeurs. Maintenant, l'élection présidentielle dépend de deux facteurs

Je voudrais tout d'abord vous donner acte, monsieur le Premier président, de votre constance. En juin 2021, la Cour des comptes a livré son analyse sur la saisine du Premier ministre. À l'époque, elle avait estimé que cette pandémie laisserait des traces durables sur l'économie française et sur les finances publiques. Vous écriviez alors : « Dans ce contexte, la soutenabilité

accru la dette publique de 560 milliards d'euros par rapport à 2019 et alourdi son poids dans le PIB de 16 points ». Vous ajoutez que « ces données situent la France dans le groupe des pays de la zone euro dont, deux ans après le début de la pandémie, la situation des finances publiques est la plus dégradée

parvenir à respecter l'objectif que le Gouvernement s'est fixé à ce jour- et encore ne s'agit-il que d'une économie par rapport à la croissance des dépenses avant-crise Cet objectif étant souvent considéré comme trop modeste, la Cour des comptes indique non sans malice, mais, bien sûr, avec la rigueur qui la caractérise, qu'il faudra « réviser l'ambition de la trajectoire des finances publiques ». Elle nous livre ensuite une quadrature du cercle, en nous rappelant qu'il faudra prendre en compte la situation économique et sanitaire, mais aussi les trajectoires de nos partenaires européens et les règles européennes en cours d'évolution- c'est là une inconnue qui ne nous invitera pas au laxisme. je fais mienne votre invitation à préciser dès le début du prochain quinquennat « les réformes nécessaires pour construire une trajectoire qui permette de garantir la soutenabilité de la dette ». Cela suppose, comme vous l'écrivez, de « faire preuve de sélectivité dans le choix des dépenses » et d'« infléchir durablement le rythme de la dépense ». Le groupe Union Centriste, s'il ne me remet pas en cause le rôle crucial de la politique du « quoi qu'il en coûte », estime néanmoins que cette politique pèsera durablement sur le déficit et la dette publique, étant rappelé que le déficit prévu en 2022 devrait atteindre le double de son niveau d'avant-crise et qu'il présente désormais un caractère exclusivement structurel. L'argent magique, on le sait, n'existe pas et les fonds déployés pendant cette crise devront être remboursés. La France se doit d'assurer la soutenabilité de sa dette pour garantir sa souveraineté et sa crédibilité. La crise sanitaire a accentué et mis en lumière les faiblesses structurelles de notre système productif, de notre modèle social et de notre

repensés ou, en tous cas, réinterrogés. Je partage ces conclusions. Claude Raynal en a dit plus sur les travaux de la commission des finances, en soulignant mon modeste rôle, et je l'en remercie. Je fais miens ses mots. La parole

nous examinons aujourd'hui le rapport public annuel de la Cour des comptes. Si ce rendez-vous est traditionnel, il n'en est pas moins essentiel pour les parlementaires que nous sommes et s'inscrit dans un contexte doublement particulier. D'une part, il permet de dresser un premier bilan des dispositifs mis en place pendant la crise sanitaire. D'autre part, il ouvre des perspectives sur les grands enjeux des politiques publiques de demain, à la veille d'une échéance électorale majeure pour notre pays. Ainsi que le rappelle la Cour des comptes, la crise a mobilisé des moyens publics importants. Cette augmentation des dépenses pèse naturellement sur le déficit et la dette publique. met en avant la nécessaire maîtrise des finances publiques, mais le redressement des comptes publics ne saurait s'entendre sous le seul prisme de la réduction drastique de la dépense. Tout d'abord, toutes les dépenses ne se valent pas et certaines sont indispensables pour préserver notre tissu économique et social, et préparer l'avenir. Ensuite, ne pas évoquer la question des recettes, alors même que les baisses d'impôts en cette fin de quinquennat ont notablement allégé les recettes fiscales, n'aurait guère de sens. Si la stratégie du « quoi qu'il en coûte » a été utile et efficace à court terme, la réaction du Gouvernement a toutefois manqué de célérité et d'ambition, sur un sujet pourtant stratégique pour l'avenir : la jeunesse. Dans un contexte économique dégradé, le Gouvernement a proposé une série de mesures en faveur de l'emploi des jeunes. De fait, le plan « 1 jeune, 1 solution », initialement doté de 6,5 milliards d'euros mais dont le coût devrait avoisiner les 10 milliards d'euros, n'a pas eu d'équivalent dans les pays comparables à la France. Pour autant, si la Cour des comptes souligne la légitimité de l'action du Gouvernement, elle regrette son manque d'efficacité eu égard aux moyens déployés. L'emploi des jeunes est certes revenu à son niveau d'avant-crise, mais la plus-value des nouveaux dispositifs n'est pas démontrée. Les mesures les plus coûteuses semblent être celles qui ont eu le moins de portée. Il en est ainsi des trois primes à l'embauche, lesquelles, pourtant, représentent 70 % des montants engagés. comptes souligne également le manque d'adéquation entre les dispositifs proposés et les besoins des publics concernés, et ce sans prise en compte des réalités territoriales. Ainsi, certains jeunes se sont retrouvés dans des dispositifs sans rapport avec leur projet professionnel, afin d'obtenir une solution financière. financière. La mise en place d'un éventail de dispositifs trop ciblés a même eu un effet contre-productif pour les publics les plus éloignés des structures d'insertion sociale. Je note, par ailleurs, que l'allocation jeunesse que nous proposions en janvier 2021 aurait pris, dans ces circonstances particulières, tout son sens. La Cour des comptes souligne en effet qu'« assurer un soutien financier à des jeunes en grande difficulté pendant la crise » aurait pu être un « objectif plus clairement énoncé », plutôt que de faire le choix de parcours d'accompagnement intensif assorti d'une allocation. La crise sanitaire a également lourdement affecté le quotidien du monde étudiant. De longues files de jeunes gens faisant la queue lors des distributions de denrées par les associations caritatives : nous avons tous vu ces images, symboles de la précarité étudiante et de la triste réalité du quotidien de nos jeunes. La Cour des comptes se comptes se montre sévère quant au soutien à la vie étudiante. Elle livre un constat sans appel sur la méconnaissance de la situation des étudiants de la part du ministère. Effectivement, comment apporter une réponse appropriée à un public que l'on ne connaît pas ? Si comparaison n'est pas raison, force est de constater que la réactivité de nos voisins européens a été plus grande. Des aides ont été versées dès le début de l'été 2020 aux étudiants les plus vulnérables ; il a fallu attendre six mois de plus pour qu'il en soit ainsi dans notre pays. De même, certains dispositifs n'ont pu atteindre leur cible. C'est le cas de l'aide à la perte d'emploi ou de stage gratifié. Cette aide de 200 euros pouvait potentiellement concerner 510 000 étudiants ; seuls 23 429 en ont bénéficié. Il faut bien dire que les critères demandés pour la percevoir ont exclu un grand nombre du dispositif. Ces critères restrictifs visaient à limiter le coût de la mesure : voilà au moins un objectif atteint La crise a mis en lumière la situation des étudiants et invite à définir des politiques de soutien à la vie étudiante adaptées : de la santé à l'insertion professionnelle, en passant par les aides du quotidien. Si nous ne partageons pas toutes les recommandations de la Cour des comptes, notamment celles qui concernent les réformes structurelles envisagées dans le cadre de la réduction des déficits publics, celles qui ont trait à la jeunesse méritent toute notre attention. La parole

comme chaque année, la présentation du rapport public annuel de la Cour des comptes est un moment important de notre vie démocratique. Ce qui me paraît préoccupant, c'est que personne ou presque ne s'inquiète vraiment de la situation de nos finances publiques. Pourtant, le rapport de la Cour des comptes met en exergue le déclassement de la France en la matière, la France devenue un facteur de risque pour la cohésion de la zone euro ! Le rapport public annuel de la Cour des comptes fait état d'un déficit structurel durablement dégradé pour la France après la crise. La Cour prône une grande rigueur d'ici à 2027 pour ramener le déficit public sous 3 % de PIB. Ce n'est pas la stratégie présentée par le Gouvernement, qui refuse la référence à une règle d'or budgétaire, pourtant plus nécessaire que jamais au regard de notre addiction à la dépense publique. On ne peut plus ni résoudre les problèmes en signant des chèques ni répondre aux conséquences de l'inflation par la dépense publique ! Ce rapport constitue tout à la fois un éclairage utile et cruel de la politique menée par l'actuel chef de l'État et un avertissement lancé à l'adresse de tous les dirigeants qui aspirent à l'Élysée. La Cour des comptes réclame un programme tout en rigueur de 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires par rapport à la trajectoire d'avant-crise pour redresser les comptes durant le prochain quinquennat. Les Allemands viennent de nous rappeler leur attachement au pacte de stabilité, alors que le gouvernement français a décidé d'envoyer sa copie seulement après les échéances ... Il existe « une divergence persistante avec nos partenaires européens », écrit la Cour des comptes, en prévenant que « cela impliquera des efforts plus importants de redressement à partir de 2023 2023- et le mur de la dette de plus en plus proche, avec une hausse inéluctable des taux qui précipitera nos finances publiques dans l'abîme -est l'année de tous les dangers. Nous sommes là ce matin pour tenter d'être des lanceurs d'alerte, dont les paroles, déjà rendues inaudibles par un « quoi qu'il en coûte » certes nécessaire, mais annihilant toute pédagogie, sont aussi couvertes, hélas, par le bruit des bottes aux portes de l'Europe. Pourtant, la Cour des comptes a su ne pas se taire et notre rôle est de faire résonner ses chiffres et les maux qu'ils recouvrent pour notre pays. Cette année, le niveau de dépenses publiques s'établira à 55,7 % du PIB, supérieur de 2 points, soit environ 50 milliards d'euros, à son niveau de 2019. Les dépenses hors crise de l'État augmenteraient fortement, de près de 11 milliards d'euros en 2021 et de 8 milliards d'euros en 2022 », écrit la Cour des comptes. Cette situation la conduit à s'inquiéter du « décalage » avec le redressement des comptes publics opéré par nos partenaires européens et à classer la France parmi les cancres de la zone euro.

élevés. » Le rapport décrit la situation réelle et inquiétante des finances publiques et met en exergue le déclassement de la France, alors que « le Gouvernement centre sa communication sur les résultats un peu meilleurs que prévu de 2021 ». Pire, ce rapport montre que malgré ce dopage à la dépense publique, nos politiques publiques sont trop souvent erratiques, inefficaces et toujours en manque d'anticipation, même sur des sujets pourtant faciles à prévoir, comme celui du grand âge, qui n'est que la conséquence de notre démographie. La Cour des comptes s'interroge en effet sur le modèle des Ehpad.

Plus largement, la question du modèle est posée et la question de son dépassement, patente. Déclassement, dépassement, redressement sont des mots si peu présents dans le débat public, quand d'autres le sont trop Les questions de l'efficacité de la dépense publique, comme de sa soutenabilité, sont clairement posées par ce rapport. C'est salutaire. La crise a pourtant montré qu'en sortant des carcans nos services publics savaient répondre aux besoins. Désormais, il nous appartient collectivement de partager ces questions, d'y apporter des réponses démocratiques pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires de notre modèle, qui est aujourd'hui dépassé et inefficace. La parole

La parole est à M. Vincent Delahaye. Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, votre rapport est excellent ! Il dresse un constat juste et, en même temps, accablant pour l'action du Gouvernement. Il alerte sur le grand déclassement de notre pays, encore aggravé par la gestion de la crise sanitaire. Hors de cette gestion de la crise sanitaire, du « quoi qu'il en coûte », les dépenses ont continué d'augmenter fortement,

Notre pays fait clairement partie des pays dits du « Club Med », ces pays du sud de l'Europe à la situation financière catastrophique. Nous sommes loin, très loin des premiers de cordée, des pays sérieux.

Il faut modifier notre fiscalité, de façon à rendre l'effort, le travail, la création et l'innovation plus attractifs. Toute baisse d'impôts doit être gagée sur une vraie

observe que la crise a révélé la précarité de certaines catégories d'étudiants, notamment les non-boursiers, insuffisamment identifiées par le ministère et par ses opérateurs. Elle ajoute que certaines mesures de soutien ont perdu en efficacité, car le ministère manquait de données suffisamment fines pour les définir correctement.

beaucoup plus simplement, fixer un cadre national précis pour l'attribution de concours financiers à la réalisation des investissements dans les Ehpad. Ce que la collégialité ne peut pas écrire, un parlementaire peut le dire. En filigrane de ces critiques, on lit les conséquences du renoncement du Gouvernement à présenter un projet de loi spécifiquement dédié à ce sujet avant la fin du quinquennat. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la loi sur le grand âge et l'autonomie

quels que soient ceux qui auront à diriger le pays. Nous avons rendez-vous avec la question des finances publiques. La Cour ne fait pas de la dette un totem ou un tabou. prône pas je ne sais quelle austérité. Elle n'est pas pour le retour à un ordre ancien, pas davantage pour un ordre nouveau. Elle souligne simplement un certain nombre de problèmes, dont l'existence est tout à fait objective,

davantage de croissance dans notre pays et, pour cela, des investissements seront nécessaires. En effet, nous avons des retards à combler. Nous avons une compétitivité à défendre et une attractivité à garantir. Nous devons investir dans la transition énergétique, dans la transition numérique,

qui sont vos interlocuteurs, de procéder désormais à des évaluations de politiques publiques locales. C'est un changement de culture, qui apportera de nouveaux éclairages sur les collectivités territoriales.

La séance est suspendue.